La deuxième série de garanties porte sur le système d'information mis en place, qui déroge au principe du secret médical

où le Gouvernement est doté de pouvoirs exceptionnels. de discussion